je rappelle que, en application de l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 août 2001 et à l'article 47 , alinéa 2, de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

même si nous aurions préféré que cette enveloppe soit fléchée vers des produits locaux et de qualité, permettant ainsi aux collectivités d'atteindre les objectifs fixés par la loi Égalim : 20 % de bio et 50 % de produits

tout en limitant les prix des repas pour les collectivités. Il s'agit d'un dispositif réclamé par les acteurs du secteur, qui prend la forme d'une prime pour le changement des pratiques et l'approvisionnement en produits locaux, bio et de qualité.

De même, on constate une baisse des prix payés aux producteurs dans certaines filières. Ainsi, certains commerces spécialisés dans la vente de produits issus de l'agriculture biologique sont actuellement en difficulté, au point parfois d'être menacés d'arrêter leur activité. Un risque de « déconversion des producteurs, qui retourneraient vers les aliments conventionnels, est pointé du doigt par les acteurs de ces filières. Pourtant, l'agriculture biologique est plus que jamais un modèle d'avenir : elle permet, outre ses bienfaits sur la santé et la biodiversité, une meilleure gestion de l'eau, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Cet élément essentiel vient nous rappeler l'importance de l'épisode de sécheresse que nous connaissons actuellement. En outre, le contexte international nous impose plus que jamais de sortir de nos dépendances : il nous faut assurer la souveraineté alimentaire des peuples et des territoires et garantir le droit à une alimentation saine et de qualité pour tous. Alors que son développement a été sous-financé ces dernières années, comme le souligne la Cour des comptes, l'État se doit de soutenir fortement la filière de l'agriculture biologique, afin de permettre au secteur de surmonter ces difficultés transitoires. de fermes bio du fait d'un manque de soutien de l'État, aggravé par la conjoncture, constituerait un non-sens historique. Dans ce contexte, et au même titre

dont l'agriculture biologique fait partie.

national des forêts (ONF) dans la gestion durable de la forêt française est essentiel, notamment pour nous préserver des conséquences du réchauffement climatique. L'ONF gère 17 millions d'hectares de forêt publique, soit 30 % de la surface forestière nationale, et assure 40 % de l'approvisionnement de la filière bois. Le Gouvernement et le conseil d'administration de l'ONF ont décidé, d'un commun accord, en juillet 2021, de supprimer 475 postes équivalents temps plein supplémentaires. Ces amendements tendent à mettre un coup d'arrêt à cette hémorragie de ressources humaines, en abondant le budget de l'ONF, afin de sauvegarder

beaucoup fait parler. En septembre 2017, le Gouvernement avait annoncé l'arrêt du financement par l'État de l'aide au maintien en agriculture biologique. Ainsi, là où les régions n'ont pas pris le relais, les agriculteurs bio

de la Cour des comptes souligne : « La question de la rétribution des services environnementaux rendus par l'agriculture bio est posée. Un tel dispositif serait de nature à renforcer la viabilité des exploitations biologiques et à inscrire leur activité dans la durée. Elle apparaît d'autant plus justifiée que les bénéfices environnementaux de l'agriculture bio profitent à l'ensemble de la société

Ils doivent en effet faire face à un changement de réglementation européenne dès 2023 nécessitant une évolution des processus d'extraction des jus, à une attaque de cécidomyies qui s'avèrent résistantes, à une pression sur les prix due à une concurrence très importante et anarchique. Les auteurs de cet amendement insistent sur la nécessité de maintenir les prix de vente de ces cultures traditionnelles, afin de permettre aux producteurs et artisans de vivre décemment de leur travail. après avoir entendu les acteurs de la filière, des mesures de proximité dédiées à une transition écologique et économique cohérente de ce secteur, qui fait la fierté de notre pays. Il s'agirait, notamment, d'encourager l'arrachage et le gel de petites surfaces de culture.

Adaptation des filières à l'évolution des marchés, du programme 149, « Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture compensée par une diminution des crédits de 10 millions d'euros de l'action n° 04, Moyens communs, du programme 215, « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Le recensement organisé par plusieurs organisations agricoles a permis d'évaluer les surfaces de serres détruites ou endommagées à 100 000 mètres carrés et d'estimer les dégâts à plusieurs millions d'euros.

leur permettre de faire face aux dégâts constatés. Ces petites fermes maraîchères diversifiées sont essentielles à notre agriculture. Elles participent à la relocalisation de notre alimentation et sont pourvoyeuses d'emplois. Quel

la promotion de la mention haute valeur environnementale (HVE), alors que ce cahier des charges est hautement contestable et contesté, et ce même après sa récente réforme, qui ne marque pas de changement en profondeur. Cette mention ne permet toujours pas de valoriser des pratiques véritablement vertueuses. Elle a d'ailleurs été votée par la Commission nationale de la certification environnementale

des mesures de soutien temporaires et exceptionnelles sont envisagées en faveur des Français, qui font face à une contraction inédite de leur pouvoir d'achat, notamment en raison de factures énergétiques largement affectées par les tensions que connaissent les marchés de l'énergie. Afin d'élargir les mesures déjà prises en faveur de l'électricité et du gaz naturel, du bouclier tarifaire, un amendement a déjà été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale dans le but de soutenir les ménages chauffés au fioul. chauffés au fioul. Or le fioul n'est pas la seule énergie à ne pas faire l'objet d'un dispositif de soutien. D'autres énergies utilisées en zone rurale, comme le bois énergie et le gaz propane, ne bénéficient d'aucun dispositif pour alléger la facture des ménages. Pourtant, les prix de l'accès à ces énergies, hors réseau de gaz naturel et en bout de réseau d'électricité, ont également connu des hausses et des aléas dans ce contexte fortement inflationniste. Il semble donc indispensable d'assurer une égalité de traitement entre les ménages : les plus précaires d'entre eux font face à des factures du même ordre

Depuis vingt ans, nous assistons à un net décrochage entre les aides personnelles au logement (APL) et les dépenses réellement supportées par les ménages. Cela s'explique principalement par des actualisations de barème insuffisantes et, surtout, par plusieurs contre-réformes menées depuis 2017, dont la plus scandaleuse restera toujours la baisse de 5 euros et la désindexation. Aujourd'hui, 77 % des allocataires supportent des niveaux de loyers supérieurs au loyer plafond des APL, alors qu'en 2001 ils n'étaient que 58 Ainsi, le Gouvernement a opéré un nombre important de coupes budgétaires sur les aides, à hauteur de 15 milliards d'euros au total, et de 4 milliards d'euros pour la seule année 2022, selon la Fondation Abbé Pierre. L'Unafo, dans une enquête sortie en 2021, a montré que la baisse généralisée des APL a surtout affecté les jeunes, avec un montant moyen diminué de 10 %. Encore une fois, comme dans toutes les crises, les jeunes payent fortement. La lutte pour le pouvoir d'achat ne peut se passer de mesures très fortes en faveur de l'aide au logement. Ce droit fondamental pèse trop lourdement sur le revenu des ménages pour que nous nous contentions des mesures actuelles. Il est nécessaire d'augmenter les aides qui bénéficient aux ménages les plus pauvres et leur permettent de mieux solvabiliser leur logement. le présent amendement, de revaloriser les APL de 10 %. Est-ce beaucoup ? Non ! C'est la simple compensation des coupes effectuées ces dernières années et le

porte sur la refacturation des dépenses d'électricité dans les résidences gérées par les communes. Les résidents des logements-foyer ne peuvent bénéficier du bouclier tarifaire de l'électricité mis en place par le Gouvernement, compte tenu de l'existence du chauffage collectif.

Dans ce contexte, les maires, ruraux en particulier, doivent pouvoir continuer à accueillir de la population dans leurs communes. La réhabilitation, la reconstruction de logements existants doivent, pour cela, être facilitées.

Pour rendre cette proposition recevable au titre de l'article 40 de la Constitution, nous l'avons financée par la diminution d'une autre ligne de la mission. Il serait souhaitable que le Gouvernement gage la création de cette nouvelle ligne par un abondement direct de 15 millions d'euros.

Cette dynamique est singulièrement préoccupante dans les grandes villes, avec l'explosion des locations de courtes durées, du type Airbnb, et l'insuffisante lutte contre l'augmentation rapide du nombre de logements vacants. certain nombre de difficultés, notamment une perte de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Afin d'orienter durablement les loyers à la baisse, nous proposons, par cet amendement, de fixer dans chaque zone un loyer de référence inférieur au loyer médian, que les propriétaires ne pourraient pas dépasser. Je le rappelle, 5 % des propriétaires possèdent 50 % des logements : ils ne sont donc pas dans l'extrême difficulté.

est ainsi libellé : La parole est à M. Antoine Lefèvre. Nous proposons d'étendre la revalorisation du point d'indice de la fonction publique aux agents salariés des 122 chambres de commerce et d'industrie réparties sur le territoire. Soumis à un statut autonome de celui des fonctionnaires, les agents publics des chambres consulaires répondent à l'obligation de respecter les principes généraux de la fonction publique. Toutefois, la valeur de leur point d'indice n'a pas connu d'augmentation depuis novembre 2010, quand celle des fonctionnaires avait été rehaussée pour la dernière fois en février 2017. Le présent amendement vise à remédier à cette situation. Si le Gouvernement a annoncé prévoir cette revalorisation par une affectation de taxe dans le PLF pour 2023,

répartis » n'ont évidemment pas vocation à abonder le budget des chambres de commerce

autant que nous sommes, nous savons qu'il est absolument nécessaire que cette transition écologique soit accélérée. Le ministre, hier, dans son intervention liminaire, a exprimé sa préférence pour les aides ciblées.

En évitant à des ménages d'être encore davantage entraînés dans la précarité énergétique, ce dispositif répond à l'urgence sociale du moment. De plus, attribué sous condition de ressources, le chèque énergie est un outil opérationnel et déjà ciblé, contrairement à certaines primes gouvernementales, pour venir en aide aux ménages les plus modestes dès l'adoption de ce texte. En complément d'une véritable politique de rénovation énergétique, qui aura des bénéfices certains à long terme, l'indexation du chèque énergie est une mesure immédiate et concrète. Quel est l'avis de la commission ? Demande de retrait. Tissot. Depuis de nombreux mois, nous assistons à l'explosion des factures énergétiques des ménages et nous constatons chaque jour, particulièrement cet été, les conséquences concrètes du dérèglement climatique. Pour répondre à ces deux enjeux, il est temps d'agir massivement sur la rénovation énergétique de l'ensemble des logements et des bâtiments privés et publics. Ainsi, nous proposons une augmentation importante du budget de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), afin de renforcer le total des aides publiques consacrées à la rénovation énergétique. Alors qu'une part très importante des crédits consacrés à MaPrimeRénov'ont été consommés et que le nombre de rénovations plafonne dangereusement, il est nécessaire de réinvestir sur cet enjeu de la rénovation énergétique. C'est une réponse de long terme, qui nous préparera à affronter de prochaines crises, mais également de court terme, avec des améliorations très rapides sur les factures énergétiques des Françaises et des Français.

l'amendement n° 278. Alors que l'urgence climatique n'a jamais été aussi prégnante, il a fallu attendre les ultimes semaines du quinquennat précédent pour que soit présenté le nouveau contrat de performance de SNCF Réseau. Ce contrat-cadre n'est ni plus ni moins que le document qui détermine les investissements sur l'ensemble du réseau ferroviaire français pour la décennie à venir. Le Sénat, par la voix de sa commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est allé jusqu'à qualifier ce document d'« occasion manquée », tant il maintient la tête de la SNCF financièrement sous l'eau, empêchant de fait une amélioration significative de l'état du réseau. Par ailleurs, Mme la Première ministre, dans sa déclaration de politique générale prononcée le 6 juillet dernier, affirmait que « le ferroviaire est et restera la colonne vertébrale d'une mobilité propre ». « Nous continuerons les investissements de ces dernières années », avait-elle ajouté. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considère que la France ne peut continuer de prendre du retard sur ses voisins européens. Il entend donc corriger cette situation, en abondant de 1 milliard d'euros le programme « Infrastructures et services de transports » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables

et notre non moins cher collègue Philippe Tabarot, vise à abonder de 1 milliard d'euros annuels les investissements ferroviaires. C'est en effet le montant qui manque, chaque année, pour assurer la régénération et la modernisation de notre réseau. Selon le gestionnaire du réseau, sans un changement de braquet dans les années à venir, nous assisterons au déclin inexorable de la performance de notre ferroviaire. On l'a dit, la signature, à l'abri des regards, pendant la campagne électorale, du nouveau contrat de performance État-SNCF

d'ajouter 1 milliard d'euros. C'est le président de l'Autorité de régulation des transports (ART) qui le dit : ce contrat de performance, pour lui, est une occasion manquée. Allons-nous oui ou non décrocher de l'Europe ferroviaire pour très longtemps ? C'est à nous d'en décider, chers collègues ! L'amendement

Depuis les années 1970, le réseau a fait l'objet de sous-investissements massifs ; il est dans un état vieillissant et dégradé. Ce contrat fait l'unanimité contre lui, que ce soit

ne porte aucune vision stratégique et industrielle, et multiplie les renoncements. C'est la raison pour laquelle, au-delà des 2,8 milliards d'euros prévus sur la régénération du réseau, l'ensemble des acteurs

ce n'est pas rien ! Il y a un besoin d'investissements massifs pour le train. Je construis actuellement, avec mes collègues du Gouvernement, le budget 2023 et la loi de programmation des finances publiques sur cinq ans. Je peux vous dire que nous aurons un vrai et beau débat sur ce sujet et qu'évidemment nous serons au rendez-vous, comme nous l'avons été depuis maintenant cinq ans.

pendant la crise sanitaire, de 4 milliards d'euros pour préserver les capacités de développement ; une enveloppe de 650 millions d'euros de crédits en faveur de la rénovation du réseau de fret ferroviaire ; et encore, je n'ai pas tout cité ! Tout cela pour dire que nous continuerons dans ce mouvement et que nous amplifierons même notre investissement pour le train.

Le fret ferroviaire a une nouvelle fois démontré sa capacité de résilience et son utilité pour assurer le transport des marchandises et l'approvisionnement des territoires. Cette activité doit être considérée comme relevant des services reconnus d'intérêt général.

vélo. La tendance des investissements actuels ne permet pas d'atteindre l'objectif fixé : voilà pourquoi nous proposons cet abondement du fonds vélo.

La dépendance aux carburants y est donc très importante : selon l'Insee, le transport est ainsi devenu le premier poste de dépenses des ménages outre-mer. Ces charges pèsent tout particulièrement sur le budget des familles modestes et des classes moyennes. C'est pourquoi cet amendement

mais, par rapport au continent, le prix du carburant affiche un différentiel moyen de 10 centimes par litre. Cet amendement vise donc à maintenir le projet initial d'indemnité carburant pour les 115 000 actifs corses qui utilisent leur voiture pour les trajets domicile-travail. Toussaint Parigi. Cet amendement vise à renforcer l'indemnité carburant pour les travailleurs de Corse, au titre de la période courant d'août à décembre 2022, afin de tenir compte de l'écart important qui existe entre le coût constaté en moyenne sur le continent et le coût, plus élevé, en Corse.

devrait prendre fin à l'automne. Son maintien et son renforcement jusqu'au 31 décembre 2022 paraissent nécessaires. Au vu de l'état des finances publiques, un tel dispositif ne pourra toutefois être prolongé de manière indifférenciée. Un dispositif de substitution ciblé, prenant en compte les professionnels « gros consommateurs », doit être envisagé. Cet amendement d'appel vise donc à attirer l'attention sur la nécessité de ne pas abandonner les transporteurs routiers, en ciblant davantage la remise à la pompe. Il tend à abonder abonder de 1 euro l'action Pilotage, support, audit et évaluations du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables », en

pour financer la dette à hauteur de 20 milliards d'euros. Bref, il s'agit d'une question de transparence. Le Parlement est là pour contrôler l'action du Gouvernement : faites-nous confiance.

monsieur le ministre

M. Vincent Segouin. L'activité des entreprises de l'événementiel professionnel français est particulièrement impactée depuis la crise du covid-19 et les nombreuses périodes de confinement. ne s'en sont pas encore remis et, en parallèle, les sites événementiels sont appelés à mettre en oeuvre des rénovations thermiques et une transition digitale qui exigent des investissements sur fonds propres, un effet de ciseaux. Cet amendement vise donc à accorder aux entreprises du secteur événementiel des instruments de quasi-fonds propres à un taux proche de l'obligation assimilable du Trésor (OAT) avec une liberté d'usage, afin d'accompagner leurs investissements pour la préparation des prochains événements qui se tiendront entre 2023 et 2025. Cette filière a vraiment besoin d'être entendue et soutenue.

Cet amendement vise à renforcer les moyens de l'Insee dans les collectivités d'outre-mer. En effet, ces territoires spécifiques manquent d'outils statistiques pour éclairer la prise de décision et le pilotage des politiques publiques. Dans une période de changements rapides comme celle que nous traversons, ces outils sont indispensables à la bonne appréciation des situations. Or, les territoires d'outre-mer ne sont pas systématiquement inclus dans les études réalisées au niveau national et ne disposent toujours pas des données nécessaires à la mise en place de politiques publiques efficaces. Quel est l'avis de la commission

établissements. Les travaux de la mission d'information du Sénat menée par nos collègues Nathalie Delattre et Jean-Marc Boyer ont montré combien la trajectoire budgétaire imposée à l'enseignement scolaire agricole était intenable.

tend à revenir sur une fragilisation du dispositif d'accompagnement personnalisé, selon laquelle une heure travaillée dans ce cadre pour les personnels correspond à une demi-heure payée. Le Gouvernement avait reconnu en 2020 que cette minoration était anormale, mais rien ne s'est passé depuis. D'autre part, il vise également à revenir sur le différentiel de rémunération important des assistants d'éducation du ministère de l'agriculture par rapport à ceux de l'éducation nationale. Cette situation d'inégalité de traitement met en difficulté les établissements agricoles. Quel Merci,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

nationale pour nos collectivités d'outre-mer. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon attendent l'issue de notre vote. Il s'agit aussi de tenir compte de la vulnérabilité particulière de nos territoires,

32 % et 24 % des familles monoparentales de Guyane et de Guadeloupe sont en situation de grande pauvreté, contre 5 % dans l'Hexagone ; la pauvreté est cinq à quinze fois plus fréquente en outre-mer qu'en métropole, en particulier dans les familles monoparentales et chez les retraités, selon une étude de l'Insee.

Mme Isabelle Briquet. L'objet de cet amendement est de permettre de revaloriser les bourses à destination des étudiants les plus démunis au niveau réel de l'inflation. Aujourd'hui, comme lors de la crise du covid-19, les étudiants et les plus jeunes subissent fortement l'augmentation des prix. L'annonce de la revalorisation des bourses à hauteur de 4 % est une bonne nouvelle dans ce contexte, mais cette hausse est inférieure au taux de l'inflation. En outre, cette revalorisation est exceptionnelle alors que les bourses devraient être indexées sur l'inflation,

et demi de plus que la revalorisation proposée par le Gouvernement. Le coût supplémentaire de cette mesure jusqu'à la fin du mois de décembre serait de 12,75 millions

Mme Raymonde Poncet Monge. Par cet amendement, fût-il d'appel, nous proposons de relever le montant de la pension minimale pour une carrière complète au niveau du SMIC.

18 % des retraités ayant une carrière complète touchent moins de 1 000 euros bruts mensuels. Pourtant, les retraites sont financées par des cotisations qui constituent du salaire socialisé. Il n'est dès lors pas normal que la pension obtenue après une vie de travail soit inférieure au niveau du SMIC.

Nous proposons donc d'augmenter le pouvoir d'achat de millions de retraités en fixant la pension minimale au niveau du salaire minimum. Il convient de garantir aux retraités des revenus décents et de leur permettre

pense, chers collègues. l'avis du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

de durée de vie. Les terribles incendies qu'a connus le pays cette année, notamment dans le département de la Gironde, ne sont que les prémices des catastrophes qui nous attendent chaque année. Le nombre de mégafeux étant amené à augmenter, il est indispensable de s'y préparer immédiatement. Si l'achat de 6 avions ces dernières années est une bonne chose, le renouvellement de la flotte de Canadair est un impératif.

le renouvellement de nos moyens nationaux, qu'il s'agisse de la flotte aérienne, du service haut débit de communications critiques, des formations militaires, de la sécurité civile ou du service de déminage.

incite à mutualiser les forces au niveau européen. À ce titre, je souhaite rappeler que grâce à l'impulsion donnée par le Président de la République lors du discours de la Sorbonne, le cadre financier européen 2021-2027 consacre 1,4 milliard d'euros à la protection civile, contre 574 millions seulement précédemment. Ce montant a donc été

la création d'une enveloppe de soutien aux projets d'investissement en matière de feux de forêt. Les auteurs de cet amendement veulent aller plus loin en proposant que l'État finance les SDIS pour opérer une campagne de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels. En plus des besoins d'investissement, une telle enveloppe de 100 millions d'euros permettrait l'indispensable recrutement d'un millier de sapeurs-pompiers professionnels. Quel

vulnérabilité face aux risques d'incendie. Il est indispensable de rapprocher les moyens de la sécurité civile des foyers de risque. C'est une demande formalisée conjointement par les présidents des départements des Landes et de la Gironde au Président de la République. La création d'une base est parfaitement compatible avec les promesses présidentielles d'étoffer la flotte de Canadair un effort européen. Il serait alors possible d'équiper cette nouvelle base dans le Sud-Ouest. Le coût de cette dernière oscille, selon les estimations, entre 16 et 18 millions d'euros. Cet amendement prévoit donc une enveloppe de 18 millions d'euros pour financer cette nouvelle base.

dès ce PLFR

à Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à prévoir la revalorisation de 10 % des aides personnelles au logement ainsi qu'à acter le principe de leur indexation sur l'inflation lorsque celle-ci dépasse l'évolution de l'indice de référence des loyers, afin que les APL ne décrochent plus,

Ils ont bénéficié aussi de la revalorisation de la prime d'activité de 4 % décidée dans ce PLFR. Ils peuvent également bénéficier des dispositifs supplémentaires qui ont été mis en place, notamment ceux que vous avez adoptés à propos des heures supplémentaires, de la monétisation des RTT et de la prime de partage de la valeur. Évidemment, nous allons continuer à les soutenir. rentrée à laquelle vous faites référence, qui a été annoncée par la Première ministre, doit, selon la copie du Gouvernement, bénéficier à 8 millions de foyers

bénéficiaires du RSA. Le sous-amendement de Philippe Mouiller prouve bien qu'il y a un vrai problème, puisqu'il faut subitement sauver les bénéficiaires de l'AAH de cette perte de 100 euros pour la rentrée ! Nous avons demandé un scrutin public, mais nous préférerions que cet amendement soit retiré purement et simplement.

Le scrutin est ouvert.

aujourd'hui, rien n'est mis en place. Il est pourtant impératif d'aboutir à un dispositif pérenne pour accompagner les ménages les plus modestes et garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous. Rappelons que 90 % des enfants et près de 70 % des adultes ne suivent pas les préconisations du programme national nutrition santé (PNNS), pour des raisons évidentes de moyens financiers. Or nous consacrons chaque année 20 milliards d'euros à soigner les pathologies cardiovasculaires et le diabète qui sont liés à cette malbouffe. L'augmentation des denrées et des

Le rapport d'enquête de 2019 montre qu'en moyenne, chaque année, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol, et 213 000 femmes déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Pourtant, seulement 18 % des femmes victimes de violences conjugales déclaraient avoir déposé une plainte en gendarmerie ou au commissariat, et 80 % de ces plaintes sont classées sans suite. En outre, le rapport de 2021 de la Fondation des femmes atteste que près de 40 % des femmes victimes de violences qui ont demandé un hébergement d'urgence, dont un tiers ayant un enfant, n'ont pas obtenu de solution. que près de 40 % des femmes victimes de violences qui ont demandé un hébergement d'urgence, dont un tiers ayant un enfant, n'ont pas obtenu de solution. Ces chiffres sont accablants, et ils nous accablent. Des ressources financières doivent être enfin dédiées à ce problème. Depuis l'année dernière, les associations estiment à 1 milliard d'euros les moyens nécessaires à la lutte contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Pourtant, le Gouvernement continue de refuser d'allouer ces moyens. Par cet amendement, nous entendons alerter quant à la banalisation des violences sexistes et sexuelles, dont la non-obtention de ces moyens témoigne.

Monge. Par le présent amendement, nous proposons d'élargir le bénéfice du Ségur social à tous les personnels des établissements de la filière socio-éducative.

des professionnels de la filière socio-éducative restent toujours écartés de la revalorisation salariale de 183 euros nets prévue dans le Ségur de la santé. En effet, les personnels techniques et administratifs des établissements de la filière socio-éducative exercent des fonctions qui sont exclues les opérateurs du 115, qui pourtant sont des rouages essentiels de l'hébergement d'urgence, ne bénéficient pas de cette revalorisation, car ils sont considérés comme des personnels administratifs, tout comme les agents d'accueil des établissements de l'aide sociale à l'enfance

Les familles font face à une augmentation élevée des dépenses : nourriture, énergie, activités extrascolaires, etc. Les fournitures scolaires ne font malheureusement pas exception. Le prix de ces fournitures va en effet augmenter de 10 % à 40 % par rapport à l'année précédente. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) stagne pendant que le prix de la rentrée explose. Revaloriser l'ARS est donc une nécessité,

est donc proposé au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » la création d'un nouveau programme « Revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire », composé d'une action unique, abondé des crédits de l'action 11 du programme 304, « Inclusion sociale et protection des personnes », à hauteur de 500 millions d'euros.

supplémentaires pour l'année 2022, de manière à répondre dès maintenant, et à les anticiper pour la fin de l'année, aux besoins de celles et ceux d'entre nous qui doivent pouvoir se nourrir- je l'espère -plus d'une fois par jour.

122 millions d'euros, et de 213 millions d'euros en 2022, soit 100 millions d'euros supplémentaires. Cette hausse est principalement portée par le déploiement du nouveau Fonds social européen (FSE) pour la période

», pour l'aide alimentaire dans les territoires ultramarins. Enfin, nous avons prolongé le dispositif Coluche prévoyant un abattement exceptionnel de 75 % de l'impôt sur le revenu pour les dons aux associations d'aide alimentaire.

En 2019, en France, 9,2 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. Ces dernières années, l'écart entre le taux de pauvreté avant et après redistribution ne cesse de se creuser, ce qui souligne le rôle majeur des prestations et des aides. Toutefois, et bien que participant largement à la réduction de 7,5 points du taux de pauvreté, les minima sociaux ne garantissent pas à toutes et tous un niveau de vie suffisant et décent.

et du logement, des sphères pourtant essentielles à l'intégration sociale. Le revenu minimum garanti consisterait en un minimum social pour chaque adulte ayant de faibles revenus,

La suppression des conditionnalités et l'automatisation du versement permettraient de réduire la pression mise sur les allocataires et de rediriger enfin les agents concernés vers leur coeur de métier, au demeurant essentiel pour retrouver un emploi : l'accompagnement, et non le contrôle.

loi de finances, tend à réviser l'indemnité de résidence des fonctionnaires, laquelle est destinée à compenser la cherté du logement. Cette indemnité de résidence a été mise en place par un décret de 1985, révisé en 2001.

la fonction publique hospitalière, est totalement insuffisante, car elle ne couvre pas l'inflation de l'année en cours et, surtout, elle ne rattrape pas le retard du gel du point d'indice des dix dernières années.

lequel nous disait : « [ ...] notre pays tient tout entier sur ces hommes et ces femmes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Il est temps de mieux les reconnaître et de mieux les rémunérer. Soutenons donc le président Macron en revalorisant le point d'indice de 10

dernières années. L'Insee confirme la hausse de l'indice glissant des prix à la consommation ; le pouvoir d'achat des Français, notamment ceux des classes populaires, s'en trouve sensiblement dégradé, les deux postes de dépense les plus touchés étant l'alimentation et l'énergie. Plus de 400 000 personnes ont basculé dans la pauvreté. Le Médiateur national de l'énergie affirme qu'un Français sur cinq a souffert du froid durant l'hiver 2021. Cette augmentation du SMIC n'est donc absolument pas superfétatoire : c'est une mesure nécessaire pour face aux dépenses essentielles, pour vivre et pour valoriser, au sens monétaire, le travail. Les cinq revalorisations automatiques du SMIC ne compensent pas l'augmentation des charges contraintes de ceux qui touchent le SMIC, et qui sont plus impactés par l'inflation. Je rappelle que ces ménages ont désépargné ou se sont endettés pour faire face au choc sanitaire et inflationniste.

Merci,

propose de reporter de deux ans la suppression du tarif réduit de l'accise sur le gazole non routier. Dans la version actuelle, le présent article ne reporte que d'un an la hausse du tarif d'accise sur le gazole non routier. Aujourd'hui, les perspectives de prix se maintiennent à un niveau très élevé sur tous les marchés de l'énergie- carburant, gaz, électricité -à court et moyen terme. Elles sont marquées par une très forte incertitude liée au contexte de la guerre en Ukraine et pourraient s'élever encore, notamment pour les carburants, compte tenu des restrictions sur les approvisionnements en provenance de Russie décidées par l'Union européenne fin mai. Il semble donc nécessaire de reporter la suppression du tarif réduit non pas d'une mais de deux années supplémentaires. Quel

Or l'inflation est réelle et nos petites entreprises ne sont pas épargnées par ses conséquences. Il est donc proposé de réévaluer le plafond d'exonération des plus-values de ces petites entreprises chaque année, au 1 janvier, en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et en arrondissant à l'euro le plus proche. La parole est à M.

en discussion commune ? Il me semble que le Gouvernement s'est engagé à ouvrir la réflexion sur les taux et les seuils applicables aux entreprises dans le cadre de la prochaine loi de finances.

L'activité de récolte de produits agricoles et leur stockage permet de bénéficier d'une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les bâtiments ruraux affectés à l'usage agricole. Toutefois, les demandes et les exigences qualitatives des consommateurs imposent de serrer et de conditionner les récoltes dans des bâtiments équipés qui permettent leur conservation, notamment les chambres froides, ce qui remet en cause cette exonération. Il est donc proposé de maintenir l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les bâtiments agricoles, indépendamment de leur caractère technique.

Aujourd'hui ne sont concernées que les communes situées en zone dite tendue, c'est-à-dire essentiellement des agglomérations. La législation actuelle exclut donc de nombreuses petites communes, notamment littorales, dans lesquelles existe pourtant un phénomène de « résidentialisation secondaire » considérable et où les prix du foncier et de l'immobilier sont bien souvent exorbitants. Mais ce phénomène se rencontre aujourd'hui partout en France. Par exemple, la commune de Paimpont, en plein Centre-Bretagne, dont j'ai rencontré le maire il y a peu,

Par ailleurs, l'amendement tend à augmenter le plafonnement de la surtaxe à 100 % au lieu de 60 % actuellement. Cette taxe est un outil important pour financer les infrastructures nécessaires aux citoyens en ciblant les ménages les plus aisés, propriétaires de résidences secondaires. Elle permet aussi de réduire la sous-occupation des logements.

nous tentons de répondre à la crise du logement dans les zones très touristiques et dans les grandes villes- comme Paris, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui en France -, en diminuant le nombre de résidences secondaires au profit des habitants. L'amendement n° 216, présenté est à M. Daniel Salmon. Cet amendement est dans la même lignée que celui que je viens de présenter. Il permet d'augmenter librement le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 % à 60 %. à 60 %. Il s'agit donc de laisser toute latitude aux exécutifs communaux, confrontés à une inflation immobilière supérieure au taux moyen d'augmentation des prix depuis dix ans- 22 % -et à un taux de résidences secondaires supérieur à la moyenne française- 13,5 % -d'augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires.

? L'avis est défavorable. Les contraintes associées aux installations éoliennes sont différentes de celles des centrales de production d'énergie photovoltaïque. Il ne nous semble pas justifié d'appliquer les mêmes règles de répartition. Par ailleurs, une telle mesure entraînerait une perte de ressources importantes pour les intercommunalités.

communale des impôts directs (CCID) rend impossible toute étude du marché locatif pour émettre des propositions de modification pertinentes en matière tarifaire ; les secteurs supposés refléter l'attractivité des loyers connaissent des variations importantes et présentent des anomalies manifestes l'échantillon statistique retenu par croisement de secteurs et de catégories est jugé insuffisant eu égard à la fixation du seuil de quatre loyers pour établir la « significativité » d'un tarif. Et encore ces remarques ne viennent que d'une commission parmi d'autres ! Pour avoir échangé avec un certain nombre

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement tend à sécuriser les projets immobiliers ayant recours à un bail à construction afin d'éviter une double taxation fiscale et de légaliser une solution administrative bien connue pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement.

du Gouvernement ? Depuis qu'il n'y a plus de conservateur des hypothèques, cette taxe finance non plus son salaire, mais la tenue par l'État du registre immobilier : elle sert donc à d'autres missions.

Je propose de mettre fin aux garanties à l'export pour les projets pétroliers et gaziers le 1janvier 2023. Cet amendement est cohérent avec la position prise par la France lors de la COP26 à Glasgow.

La suppression de l'ISF n'a eu aucun effet sur l'investissement. Cette mesure s'est finalement réduite à la mise en place d'un dispositif qui a un peu plus enrichi les contribuables les plus aisés, ceux dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Comme l'indique Oxfam, le patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50 % de la population. Or ces gaz à effet de serre posent problème. Nous proposons donc un outil de justice climatique. Notre amendement vise à introduire, par rapport à l'ancien ISF, un nouveau barème d'imposition associé à des taux plus progressifs

d'euros. Les propriétaires appartenant à la classe moyenne sont concernés par cet impôt, compte tenu de la flambée des prix immobiliers. En effet, 20 % des Français qui paient l'IFI ont des revenus inférieurs à 5 000 euros par mois.

observer des disparités territoriales importantes. Seules trois régions ont enregistré une baisse du prix de l'immobilier en 2021 : les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et l'Île-de-France, hors Paris. En revanche, d'autres régions ont connu une nette augmentation.

Conséquence : de nombreux contribuables considérés comme des classes moyennes supérieures ne pourraient plus aujourd'hui acheter le logement qu'ils occupent depuis des années. Certains sont même contraints de déménager. Aussi, je vous propose

La hausse des prix du carburant affecte directement le pouvoir d'achat des 6 millions de Français vivant en zone de montagne, qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou pour accéder

L'objectif est avant tout d'appeler l'attention du Gouvernement sur la situation de l'île. Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de la Corse dès à présent, afin de pouvoir proposer des dispositifs plus ciblés dans le budget pour

La hausse du prix des carburants affecte directement le pouvoir d'achat de millions de Français, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre au travail ou accéder aux services

restructurer leur dette a souvent comme conséquence de dégrader leur notation à la Banque de France, raison pour laquelle peu d'entre elles se sont emparées de ce dispositif. Pourriez-vous m'indiquer les démarches que vous comptez entreprendre pour leur ménager un allongement de remboursement de ces prêts

Anglars, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié. Cet amendement vise à accorder aux habitants des communes classées en zone de montagne une déduction forfaitaire supplémentaire de 5 % sur leurs revenus, prenant en compte les surcoûts que représentent les coûts de l'énergie dans les territoires de montagne.

paraît complexe, sachant que les communes situées en zone de montagne représentent 18 % du territoire national et qu'elles ne sont pas, loin

même parfois subvenir à leurs besoins. L'article 156 du code général des impôts définit le revenu imposable et les sommes qui peuvent en être déduites sous certaines conditions. Aujourd'hui, parmi les aidants, seuls les obligés alimentaires- ascendants ou descendants directs -peuvent bénéficier de ce dispositif. Cet amendement Cet amendement a donc pour objet de déduire du revenu imposable les sommes versées par tout proche aidant, afin de leur permettre de bénéficier de ce dispositif fiscal, en plafonnant la part des charges susceptibles de faire l'objet d'une déduction d'impôt à 30 % des revenus du proche aidant.

temps, énergie et ressources à des activités allant dans le sens de l'intérêt général.

de publier dans les six mois un bilan carbone renforcé et standardisé, une stratégie climat et un plan d'investissement permettant de mettre en oeuvre cette stratégie.

Les établissements hospitaliers de Corse ne sont actuellement pas en mesure de proposer aux patients qu'ils accueillent tous les traitements que nécessite leur état de santé. Ces carences s'illustrent, par exemple, par l'obligation de disposer d'un recours aux équipements continentaux de niveau 3 et, pour certaines spécialités chirurgicales et médicales, par la nécessité de garantir

et 108 du traité, les aides à l'investissement à finalité régionale ne peuvent concerner que des aides à finalité régionale octroyées pour un investissement initial, ce qui n'est pas forcément le cas des aides mentionnées dans le présent

? Ce transfert est effectif depuis le 1 janvier 2022. Il s'inscrit dans le mouvement d'unification du recouvrement,

et en faire un instrument de lutte contre l'urgence climatique. Elle permettrait de fixer les règles d'une fiscalité écologique plus juste, plus efficace, plus incitative que punitive, plus cohérente et plus protectrice pour les Français. Ces conditions sont un prérequis indispensable pour pouvoir évoquer une nouvelle trajectoire pour la fiscalité écologique, qui est indispensable au regard de l'urgence climatique.

finances pour 2021 de conférer une garantie de l'État à un projet immobilier d'un établissement scolaire français à l'étranger. Cet amendement tend à élargir cette possibilité non seulement aux établissements, mais aussi à des entités juridiques qui seraient dédiées au développement d'un projet immobilier. Un tel assouplissement est nécessaire dans certains pays, compte tenu des statuts des établissements scolaires et de la manière d'optimiser les projets immobiliers. projets immobiliers. Nous pourrions ainsi ouvrir la possibilité de garantie de l'État à des véhicules juridiques spécifiques qui opèrent un projet immobilier pour le compte d'un établissement en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Cette mesure est indispensable pour permettre le développement du réseau.

est défavorable. Le dispositif serait inopérant : ces établissements font partie intégrante de l'AEFE qui est soumise à la règle de non-endettement des organismes divers d'administration centrale (ODAC)

Olivier Cadic, pour explication de vote. Techniquement, ces amendements reviennent à offrir à un établissement public, en l'occurrence l'AEFE, les moyens de contourner l'interdiction d'emprunter, sans aucun contrôle de la représentation nationale. nationale. Il est donc proposé qu'une agence d'État puisse créer des structures juridiques à l'étranger pour faire des emprunts immobiliers en faveur de ses 67 établissements en gestion directe. Utiliser Utiliser le PLFR pour faire avancer de tels mécanismes a de quoi surprendre : je ne voterai donc pas ces amendements. Je mets aux voix

à une alimentation de qualité- nous avons déjà eu l'occasion de le signaler. La restauration scolaire joue, à cet égard, un rôle essentiel pour les familles défavorisées. Or, cela a été dit, les collectivités font face à l'inflation des prix alimentaires. Certaines d'entre elles pourraient être contraintes d'augmenter leurs tarifs. cette raison, cet amendement a pour objet d'étudier, à travers un rapport, la mise en place du financement par l'État de la généralisation de la tarification sociale de la restauration scolaire.

échéant applicable. Sans remettre en cause la généralisation de l'utilisation de factures électroniques par tous les acteurs économiques ni le calendrier de cette réforme, cet amendement vise à prendre en compte les capacités des plus petites entreprises et un risque élevé d'erreurs de leur part. Toutes ne seront pas prêtes en 2026. Le présent amendement a pour objet de réduire le montant de l'amende par facture à 5 euros et celui de l'amende par transmission à 50 euros, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 5 000 euros.

bis La parole est à M. Antoine Lefèvre, sur l'article. J'ai souhaité prendre la parole sur cet article, car il m'a paru important de rappeler quelques-unes des nombreuses initiatives que notre chambre a prises au cours des dernières années en faveur des Américains dits accidentels, ces Français devenus américains par leur naissance sur le sol des États-Unis.

Le 14 février 2022, les huit présidents de groupe parlementaire du Sénat se sont associés pour adresser au ministre de l'économie un courrier, visant à l'encourager à profiter de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE) pour porter le sujet à l'échelle européenne et faire avancer les négociations avec l'administration américaine.

Toutefois, l'immobilisme auquel doivent faire face ces Américains accidentels depuis plus de huit ans exige que des actions fermes soient engagées dans les plus brefs délais. Pour cette raison, je voterai le maintien du dispositif tel que proposé par l'amendement d'Olivier Marleix à l'Assemblée nationale. Je ne voterai pas l'amendement de suppression proposé par le rapporteur général.

L'important, pour le moment, est de pouvoir actionner les leviers qui sont à notre disposition et de sortir, dans les meilleurs délais, les Américains accidentels de cette situation kafkaïenne. Un vote conforme à celui de l'Assemblée nationale montrera une unité et une détermination du Parlement français dans la volonté de renégocier les clauses de l'accord Fatca. Il poussera le Gouvernement à se montrer plus déterminé dans ses tractations avec Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain. Il faudra au premier chef examiner la possibilité de négocier l'établissement d'une procédure facilitée

Il a été ratifié par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2014. La Constitution française prévoit expressément à son article 55 la primauté du droit international sur le droit interne. Selon le droit américain, toute personne née sur le sol américain est citoyen américain

Le dispositif tel que rédigé par le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale voudrait imposer une réciprocité pour appliquer le traité. Il signifie pour les Français des États-Unis qu'ils devraient déclarer leurs revenus américains en France et, éventuellement, payer des impôts en France sur ces revenus. Cela contreviendrait à la convention fiscale bilatérale et à tous nos principes et exposerait les établissements financiers français à des sanctions américaines, s'ils ne respectaient pas l'accord. Je voterai l'amendement du rapporteur général, qui élimine à la fois ces risques et un dispositif qui ne réglera en rien la situation des Américains accidentels, en plus d'être inconstitutionnel.

des difficultés rencontrées par les Américains accidentels. Le processus de renoncement à la citoyenneté américaine est entièrement entre les mains de l'administration des États-Unis, et ce quelles que soient les conditions d'application de la loi Fatca.

sans rapport avec les obligations fiscales, qui, en France, sont basées sur la territorialité de l'impôt, mais cela entretiendrait aussi l'incompréhension de nos ressortissants, créant un précédent fort préjudiciable pour l'ensemble des Français établis à travers le monde. Cet article 10 ne règle pas le problème de fond de la débancarisation des Américains accidentels et des Français vivant aux États-Unis. La politique systématique de la part des banques françaises, les seules en Europe à pratiquer ainsi à grande échelle, est de clore les comptes de nos ressortissants

d'intérêt que j'ai été l'auteure de l'amendement qui avait introduit le droit au compte bancaire dans le droit français en 2011.

l'amendement n° 114 rectifié. Selon qu'un justiciable est une personne morale ou un particulier, il est soumis à un traitement fiscal différent, ce qui est de nature à créer des inégalités dans l'accès au droit et à la justice, notamment dans l'aide juridictionnelle. Cet amendement vise à mettre en place une aide qui prendrait la forme d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt serait fondé sur le même mécanisme que celui existant en matière d'emploi d'un salarié à domicile. Il serait pris en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux ; s'il excédait l'impôt dû, l'excédent serait restituable. restituable. Les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt qui seraient déjà prises en compte pour l'évaluation des revenus imposables d'un contribuable ou qui seraient prises en charge par l'aide juridictionnelle n'ouvriraient pas droit à ce dispositif. Ce crédit d'impôt permettrait ainsi de réduire cette inégalité injustifiée entre les particuliers et les entreprises selon leur statut fiscal, tout en améliorant l'accès au droit pour les foyers modestes.

plusieurs années : l'article 568 du code général des impôts qui définit le nombre de licences de vente du tabac accordées dans les départements d'outre-mer, qui résulte de l'article 134 de la loi 2011-1977 de finances du 28 décembre 2011 pour 2012 et qui nécessitait un décret d'application n'ayant jamais été pris

Si 671 prêts ont été décaissés depuis 2020, on constate un fort tarissement des flux de demandes depuis le second semestre 2021. Cette tendance s'est encore renforcée en 2022, ce qui montre l'épuisement du vivier des entreprises éligibles à ce dispositif. À des fins de clarté et de rationalisation des dispositifs d'aide aux entreprises, il est pertinent de ne pas prolonger le dispositif spécifique des prêts participatifs, tout en maintenant les prêts garantis par l'État et les prêts bonifiés pour les entreprises touchées par les conséquences de la guerre en Ukraine.

M. Daniel Salmon. Cet amendement prévoit de supprimer le caractère rétroactif de la mesure prévue à l'article 13. La rétroactivité affecte la crédibilité du soutien public aux énergies renouvelables en France. Les investisseurs pourraient se détourner de ce secteur et les banques durcir leurs conditions de financement.

Cet amendement prévoit que les modalités de cet arrêté soient établies en concertation avec les acteurs de la filière des énergies renouvelables, afin qu'ils puissent faire part de leurs situations particulières. Il convient ici de le rappeler, les énergies renouvelables, le mécanisme qui régit leur intégration au marché de l'énergie, permettent de générer des recettes nouvelles pour l'État à un moment où il est nécessaire de mobiliser des fonds pour soutenir le pouvoir d'achat des Français.

de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité de 2011 faisait un premier état des taxes, exonérations et subventions qu'il conviendrait de réviser ou supprimer. Nombre de ces outils fiscaux existent encore aujourd'hui, et parmi eux l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes ou encore les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Cet abattement n'a pas de sens. C'est pourquoi cet amendement vise à le supprimer et à le limiter aux parkings couverts par des panneaux photovoltaïques afin d'inciter au développement des énergies renouvelables nécessaires à notre souveraineté énergétique.

ruraux alimentés au minimum à 70 % par des énergies renouvelables ou de récupération, en permettant aux collectivités de les exonérer de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises. Quel est l'avis de la commission ? Demande de retrait.

Nos consulats ont déjà délivré cette année plus de titres sécurisés que pendant toute l'année 2019. Ils n'en peuvent plus et ont besoin de moyens. Cet amendement est un appel à la solidarité, monsieur le ministre, un appel

renforcerait le soutien aux projets d'investissement des communes et, surtout, permettrait de consommer la totalité de l'enveloppe et de ne perdre ni les projets ni la subvention DETR. Quel est l'avis de la commission ? J'ai le sentiment

demande est satisfaite à droit constant, puisqu'une souplesse a d'ores et déjà été donnée aux préfets par le décret du 8 avril 2020 qui leur permet de déroger aux articles réglementaires relatifs aux subventions attribuées aux collectivités locales, lorsque cela est justifié par des circonstances locales et pour des motifs d'intérêt général.

en fonction de strates de collectivités- régions, départements, communautés de communes, syndicats, communes, etc. -, un certain nombre de différences. J'avais conçu cet amendement comme un amendement de repli par rapport à celui qui a été très largement adopté tout à l'heure par le Sénat. Quoi qu'il en soit, ces informations nous seraient utiles. Je suis soucieux de savoir ce que le Gouvernement souhaite faire,

Ils sont liés à l'application des décrets issus du Ségur de la santé, qui revalorisent les primes de certains personnels relevant de la fonction publique territoriale.

Défavorable.

Le Gouvernement souhaite rappeler pour coordination l'article d'équilibre, à savoir l'article 5 et l'état A, pour tirer les conséquences des votes intervenus lors de l'examen de la seconde partie du texte. seconde partie du texte. En application de l'article 47 , alinéa 3, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une coordination de l'article d'équilibre, article 5 et état A, du projet de loi de finances rectificative pour 2022.

remet à la sagesse du Sénat. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.